Madame la présidente,

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, le sport transcende les clivages, y compris dans cet hémicycle. Sa portée universelle nous permet, un temps, de mettre de côté nos différends. Son utilité sociale n'est plus à démontrer. Alors que de plus en plus de personnes s'inquiètent d'un délitement de la société, il fait partie de ces outils essentiels à la République émancipatrice que nous souhaitons. C'est d'autant plus vrai qu'il permet souvent aux populations les plus fragiles socialement et économiquement de sortir la tête de l'eau et d'échapper aux difficultés du quotidien. Il n'est d'ailleurs pas étonnant que l'on constate, en même temps que la fermeture des lieux sportifs, une augmentation de 80 % des troubles d'ordre psychologique chez les jeunes de moins de 15 ans. Il y a encore peu, la France s'était donné comme cap d'accueillir les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 avec une progression de trois millions de pratiquants sportifs. Sans même entrer dans le débat autour de la dénomination de ces pratiquants, la pandémie nous oblige à revoir nos plans. Aujourd'hui, ce sont 180 000 clubs et 108 fédérations qui sont en souffrance. Clubs de danse, de gymnastique, d'arts martiaux, de basketball, de rugby, etc. : plus de 70 000 structures craignent de ne jamais pouvoir rouvrir.

Ce constat est d'autant plus accablant qu'il existe de fortes disparités selon les territoires et les disciplines. J'étais lundi dernier dans les quartiers nord de Marseille, ma commune, au comité de veille de La Busserine. Là-bas, 65 % des licenciés ne sont pas revenus, alors même que le confinement a été particulièrement éprouvant pour eux et que la pratique libre du sport n'est plus possible. Pire, la fermeture des locaux a entraîné une occupation des lieux par des dealers. Or les bénévoles ne savent pas s'ils pourront les les faire partir une fois l'activité sportive relancée. À cela, il faut ajouter près de 120 millions d'euros de pertes de recettes issues des événements et du sponsoring. Je salue l'engagement

Face à cette situation cataclysmique, les pouvoirs publics doivent être en mesure de répondre à trois questions. Qu'a-t-il été fait jusqu'à présent ? Quelles réponses apporter dans les semaines et les mois qui viennent ? Quelles leçons tirer de la situation ? Madame la ministre, je ne doute pas un seul instant de votre attachement à la pratique sportive, qui fait votre quotidien depuis tant d'années. Force est toutefois de reconnaître que, jusqu'à présent, les réponses à la crise de votre ministre de tutelle et du Gouvernement ne sont pas satisfaisantes. J'y vois d'ailleurs un nouvel effet indésirable du rattachement forcé de votre ministère à celui de Jean-Michel Blanquer.

Voilà, en substance, la réponse apportée pour le gros des associations sportives. Pour être tout à fait exhaustif, il faut citer également l'accompagnement des 30 000 associations sportives employeuses, qui peuvent bénéficier du chômage partiel et des prêts garantis par l'État

où il y a de gros intérêts en jeu. Celui-là, il est visiblement plus important que les autres, on ne l'a pas sacrifié. L'économie prime sur tout, on l'a tous bien compris. » Bien sûr, les pertes à assumer pour le sport professionnel, ainsi que sa place dans le paysage économique du pays, sont d'un tout autre Les chiffres sont connus : des pertes de recettes dépassant allègrement le milliard d'euros, près de 350 000 emplois directs concernés et plusieurs milliards d'euros de retombées fiscales en temps normal.

Même en matière sportive, on ressent une sorte de « deux poids, deux mesures » qui interroge. À ce titre, est-il pertinent d'avoir relancé et maintenu avec tant d'ardeur les compétitions professionnelles, tout en laissant au placard les compétitions amatrices

Malgré cette proximité, et les échanges entre les trois villes, un seul des trois clubs est interdit de compétitions, alors que les protocoles sanitaires sont appliqués partout. C'est d'autant plus incompréhensible

La mise sur le marché la semaine dernière du masque fabriqué par Salomon peut-elle constituer une porte de sortie de crise pour les associations sportives ? Si oui, votre ministère s'engagera-t-il financièrement et matériellement pour aider les fédérations et les clubs à se doter en matériel ? De façon moins immédiate, cette crise montre que notre modèle sportif a atteint ses limites. On pourrait presque se poser la question : le sport professionnel est-il devenu fou ? Le sportif et le supporter que je suis est parfois

encore, certains clubs exprimaient leur volonté de renforcer leur indépendance vis-à-vis de l'État, tout en attendant de ce dernier un soutien financier important. On en revient à la privatisation des profits et à la mutualisation des pertes, qui prévaut déjà dans la gestion des stades.

grandement en difficulté le football professionnel, a une conséquence que l'on évoque trop peu souvent : il prive toutes les disciplines sportives amatrices d'une manne essentielle à leur survie. Depuis plusieurs années, des économistes pointent le risque d'implosion de la bulle des droits télévisés et de celle des transferts, mais aussi le problème de l'endettement des clubs, et appellent à revoir le modèle sportif professionnel. Il me semble qu'un chantier devrait être lancé autour du plafonnement des taxes liées au sport. Selon les documents budgétaires présentés par le Gouvernement, les taxes sur les paris sportifs, les jeux de loterie et la taxe Buffet représenteront en 2021 une recette d'environ 420 millions d'euros, pour un reversement à l'ANS estimé

Toutefois, je me joins à la colère de ma collègue Marie-George Buffet qui, me semble-t-il, a une certaine légitimité en matière sportive. Comment démocratiser le sport sans avancer sur le dossier de la régulation du monde professionnel, tout à la fois apporte les moyens nécessaires au monde amateur, mais capte une part non négligeable des ressources publiques ? Comment démocratiser le sport sans s'atteler à la question de l'engagement de l'État dans la pratique sportive, alors même que votre ministère ne représente que 0,14 % du budget de l'État ? Comment démocratiser le sport sans évoquer la question du sport scolaire, qui constitue un outil essentiel à l'épanouissement des enfants comme une porte d'entrée à la pratique licenciée ? Comment, enfin, démocratiser le sport sans s'atteler à tous les freins à la pratique, notamment économiques ? En cette période de crise, les sports amateurs et professionnels ressemblent de plus en plus à un champ de ruines. Si la situation est catastrophique, elle offre aussi l'opportunité de repartir sur de bonnes bases. Ce débat, qui préfigure d'une certaine manière la discussion sénatoriale sur la proposition de loi de Céline Calvez, doit être l'occasion de proposer des solutions pour un avenir sportif populaire

M. Claude Kern. Madame la ministre, il y a trois semaines, vous nous annonciez une bien mauvaise nouvelle. La reprise du sport amateur au sens large n'aura pas lieu avant plusieurs semaines, certainement pas à Pâques, compte tenu du presque reconfinement, peut-être à la Trinité, voire aux calendes grecques- ironie du sport à la veille des jeux Olympiques, dont il n'est certes pas question ici, quoique Pas plus tard que ce week-end, plusieurs fédérations ont en effet déjà annoncé l'arrêt du sport amateur pour cette saison. Or c'est bien une pratique sportive, populaire et accessible à tous, en d'autres termes la reprise d'une activité essentielle en termes de santé physique, d'hygiène mentale,

Il est heureux que le plan de relance décidé à l'automne dernier ouvre des perspectives, là où le sport figurait dans l'angle mort du déconfinement et du retour vers une vie en société. ne sommes pas seulement dans l'insuffisance moribonde, nous sommes dans la suffisance d'une majorité gargarisée par de belles paroles qui n'engagent à rien quand elles ne sont pas confrontées à la réalité. Certes, de nombreux efforts ont été accomplis en complément des aides de droit commun déjà mises en place par le Gouvernement Fonds d'urgence pour les fédérations sportives, Pass'Sport, Fonds de compensation de pertes de billetterie, etc. En l'espèce, dans un souci d'exigence et c'est désormais une préoccupation d'urgence,

Aussi, alors qu'un pan entier du socle de nos valeurs communes est en train de s'effondrer, qu'en est-il concrètement de votre projet à leur endroit ? « Le réel, c'est quand on se cogne », n'est-ce pas ? Madame la ministre, quelles nouvelles alarmes de santé publique faudra-t-il

On le sait, la sédentarité et l'inactivité prolongée ne sont pas qu'un spectre fantasmé aux contrecoups hypothétiques : c'est une entaille profonde et attestée dans l'idée même de santé publique, dont les conséquences sont trop bien déterminées. Les plus jeunes sont en première ligne

à l'échelle d'un petit d'homme ou d'un jeune citoyen à l'esprit sain dans un corps sain ? de votre volonté, de votre agenda, des moyens, et pas seulement pour les trois prochaines semaines Qu'en sera-t-il de la mise en oeuvre du plan 2020 et de ses belles idées, « véritable enjeu de santé, d'épanouissement, d'égalité et de réussite pour les élèves », selon vos propres mots ? la ministre, comment comptez-vous dépasser l'horizon funeste et pénible de la sédentarité et de la perspective d'anomie. Quel est votre projet au-delà d'un sport pour la jeunesse enfin ressuscitée ?

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, je commencerai par féliciter nos collègues du groupe CRCE d'être à l'origine de ce débat auquel la conjoncture actuelle apporte un écho démultiplié. Ne nous berçons pas d'illusions, le sport sortira sérieusement affaibli de la crise sanitaire : le nombre de licenciés aura régressé dans des proportions inquiétantes ; des bénévoles resteront à la maison ; des clubs amateurs disparaîtront ; des structures professionnelles connaîtront une adaptation difficile ; certains événements auront du mal à renaître. Les loisirs sportifs marchands enregistrent d'ores et déjà des pertes financières considérables. Par exemple, l'Union Sport & Cycle annonce une perte de 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires cette saison pour les commerces et fournisseurs d'équipements de ski. Bref, tout l'écosystème sportif se trouve affecté par une crise inédite. Dans ce contexte, je salue les efforts déployés par Mme la ministre et ses services, ainsi que par les fédérations, notamment afin de proposer des protocoles sanitaires adaptés à chaque situation. Rendre l'activité physique accessible au plus grand nombre justifie l'existence d'un service public du sport, qui est un bien collectif à partager. En d'autres termes, la promotion d'un authentique sport pour tous nécessite une politique publique affirmée et globale, en phase avec les évolutions contemporaines. Pour donner de la respiration financière aux clubs sportifs, au moins trois mesures exceptionnelles doivent être envisagées jusqu'à l'été 2024 : d'abord, rehausser de 60 % à 80 % le plafond de réduction fiscale des dons aux associations sportives pour encourager le mécénat transformer une partie du coût des adhésions et licences en dons donnant lieu à crédit d'impôt pour réduire l'hémorragie du nombre d'adhérents ; enfin, relever le plafond des taxes affectées au financement de l'Agence nationale du sport.

Une enquête réalisée par l'Association européenne des professeurs d'éducation physique et sportive montre que 40 % des élèves présentent une augmentation de leur masse graisseuse et une diminution de 16 % de leurs capacités aérobies. Les tests réalisés à l'issue du premier confinement indiquent une perte de capacité physique des élèves de CE2 de l'ordre de 20 %. La proposition de loi débattue la semaine dernière à l'Assemblée nationale aurait pu être l'occasion de redonner ses lettres de noblesse à l'éducation physique et sportive. Le rapprochement ministériel entre l'éducation nationale et le sport restera de l'ordre du symbole tant que ne sera pas augmenté le nombre d'heures d'EPS de la maternelle à l'université et qu'un continuum sport éducatif-sport fédéral ne sera pas effectif.

Il est urgent de doter les politiques sportives d'un financement durable reposant équitablement sur le rendement financier produit par l'activité sportive elle-même, d'où le slogan : « Le sport doit financer le sport !

physiques et sportives (APS) en renforçant l'accompagnement du public spécifique et en assurant l'égalité d'accès aux pratiques est un enjeu majeur. Des efforts doivent ainsi être conduits pour promouvoir la mixité dans l'éducation sportive et pour lutter plus efficacement contre le sexisme et l'exclusion dont font l'objet les jeunes filles et les femmes dans l'exercice d'activités, dont l'offre n'est pas toujours adaptée et suffisamment diversifiée. Une plus grande inclusion et une meilleure accessibilité des personnes en situation de handicap constituent également un objectif vers lequel nous devons tendre en modernisant les équipements et en développant des politiques plus ambitieuses de promotion du handisport. d'un sous-investissement chronique et persistant, l'état de notre parc d'équipements sportifs, y compris scolaire, doit faire l'objet d'un plan global de modernisation. Le problème se pose, en particulier, pour les piscines, qui n'ont pas fait l'objet de financement d'envergure depuis le grand plan d'équipement lancé en 1971. Depuis de nombreuses années, lors de chaque débat budgétaire est rappelée l'urgence de lancer un ambitieux plan de rénovation-construction d'installations et équipements, avec une recherche de mixité des usages, pour que puissent y cohabiter des sportifs pratiquant dans un cadre institutionnel, mais aussi des personnes venues pratiquer une activité de loisir. La montée en puissance des exigences environnementales et territoriales est à intégrer, au-delà de la prise en compte impérative des zones dites carencées, notamment les quartiers prioritaires de la politique de la ville et les zones de revitalisation rurale La problématique d'une pratique sportive populaire et accessible à tous pose la question du droit au sport. Depuis les années 1980, nous connaissons une croissance des activités autonomes dans l'espace public, des pratiques libres ou encadrées dans des structures commerciales.

Les inégalités territoriales, socioculturelles, économiques, genrées demeurent élevées. À l'aune de la réduction de ces inégalités, la gestion de l'après-covid représentera une période test pour la nouvelle gouvernance du sport français, pour le rôle de l'ANS et de ses déclinaisons territoriales. En effet, les conférences régionales du sport et les conférences des financeurs, qui se mettent progressivement en place sur le terrain, ont pour mission d'associer plus étroitement l'ensemble des acteurs susceptibles de contribuer au développement de l'offre d'activités physiques et sportives parcours sportif des enfants, pratique des populations adultes dans leur diversité, etc. L'intitulé de notre débat de ce soir rappelle l'importance du sport de masse ou du sport pour tous. Il sous-entend que l'accès au sport doit être considéré comme un droit,

des exigences éminemment concrètes : assurer un accès pour tous aux équipements, favoriser un développement équilibré des pratiques sur l'ensemble du territoire national et tout au long de la vie, diversifier les métiers de l'accompagnement sportif. Sur ce dernier point, les chiffres de Parcoursup parlent d'eux-mêmes : aucun autre secteur de recrutement ne connaît une telle saturation en matière d'orientation. Aussi le moment est-il sans doute venu de conduire une réflexion sur une nouvelle diversification des métiers du sport. En matière d'encadrement, le recul de 80 % en trois ans des emplois aidés du secteur associatif est fortement préjudiciable à son dynamisme. Le rebond de la pratique passe par une relance de l'emploi sportif qualifié dans les clubs, lesquels demeurent la cellule de base institutionnelle dans un univers de pratiques différenciées. Ces structures doivent se penser comme étant au centre d'une articulation de tout un ensemble de pratiques publiques : sport et éducation, sport et santé, sport et entreprise, sport et développement économique, sport et aménagement du territoire, sport et environnement, sport et tourisme, sport et réinsertion sociale, etc. Au coeur de cette transversalité se distingue une

Au-delà des mesures d'urgence, le sport français a besoin d'un nouveau cadre et d'objectifs réactualisés. La proposition de loi visant à démocratiser le sport en France a commencé à tracer des perspectives. Les réactions qui ont suivi son adoption sont révélatrices de manques qu'il reste à combler. Un quotidien du soir titrait hier : « La proposition de loi sur le sport provoque frustration et regrets. » Puisse l'examen prochain de ce texte au Sénat contribuer à donner contenu et rayonnement au titre ambitieux qui est le sien. La première priorité d'une politique sportive nationale doit être de développer le nombre de pratiquants, ce qui suppose une forte capacité d'action de la part de l'État, avec un ministère doté de moyens financiers supplémentaires, à un moment où le sport français est en danger. Par ailleurs, n'oublions pas qu'il peut fortement contribuer à renforcer la cohésion sociale et éviter les dérives populistes menaçant notre société. L'héritage olympique était censé amener une augmentation de 10 % du nombre de pratiquants en 2024, un objectif exprimé par le Président de la République. Ayons le courage de dire que cette ambition est devenue caduque. Notre intention de court terme est plutôt de retrouver la situation d'avant-covid. Depuis un an, nous n'avons jamais autant entendu parler de facteurs de comorbidité, mais également de l'apport de l'activité physique pour faire face à ces facteurs, dans le domaine tant préventif que curatif. Cette réalité doit nous encourager à poursuivre collectivement ce combat pour le développement de la pratique sportive. Je termine sur ce message d'espoir, qui doit susciter une meilleure prise en compte du sport dans notre société et, plus largement, du corps dans notre vie.

Depuis plus d'un an, une crise sanitaire sans précédent s'est abattue sur notre pays. Depuis plus d'un an, nos espaces de vie sociale sont profondément modifiés : nombre d'activités sont à l'arrêt, l'activité physique et sportive ne faisant malheureusement pas figure d'exception. Durant le premier confinement, 38 % des Français ont diminué leur pratique sportive. Ce chiffre est loin d'être négligeable, même si, sur l'année 2020, la part de pratiquants reste relativement stable, puisque 65 % des Français ont pratiqué au moins une activité sportive dans l'année écoulée, contre 66 % en 2018. Il convient également de souligner que, durant ce premier confinement, contrairement aux idées reçues, quasiment aucun non-pratiquant ne s'est mis à la pratique sportive. Le secteur du sport amateur en club et association a lui aussi connu un coup d'arrêt brutal. Après la stupeur des premiers instants, les acteurs ont tout fait pour organiser une reprise dans les meilleures conditions. Las, depuis un an, la pratique en club n'a été autorisée que durant quelques semaines entre les mois

ces structures ont pu accéder aux dispositifs de droit commun, mais il est regrettable qu'aucun véritable plan ambitieux pour le sport n'ait été présenté à ce jour pour bien préparer la reprise. Les pertes financières sont là et elles seront très difficiles à surmonter. de vue humain, de nombreux clubs craignent aussi de souffrir d'un désengagement des bénévoles, qui sont pourtant la ressource clé de la majorité de ces structures.

Afin d'assurer une reprise de la pratique sportive populaire et accessible à tous, le Président de la République a annoncé, au mois de novembre dernier, la création d'un Pass'Sport, à hauteur de 100 millions d'euros. Si nous pouvons saluer cette idée, de nombreuses questions restent malheureusement en suspens, et j'espère que nous pourrons avoir des réponses ce soir.

Qui pourra en bénéficier ? Sous quelle forme et pour quel montant ? Il est également regrettable que ce Pass'Sport ne soit pas universel, à l'instar du Pass'Culture. Encore une fois, cela souligne malheureusement la différence de traitement entre le sport et la culture. Un autre moyen de soutenir la reprise sportive serait de permettre aux licenciés et adhérents des salles de sport de voir leur adhésion considérée comme un don ouvrant droit à une défiscalisation. Cette Cette proposition aurait le mérite de bénéficier à un public différent de celui qui sera concerné par le Pass'Sport, étant donné que celui-ci serait soumis à des conditions de ressources. Madame la ministre, que pensez-vous d'une telle initiative ? Je tiens à rappeler que de nombreux pratiquants en club comme dans les salles de sport privées ont pris leur licence ou leur adhésion lors de la rentrée 2020. Depuis, la plupart d'entre eux n'ont quasiment jamais pu pratiquer dans ce cadre et beaucoup se posent la question de la rentrée Si certaines fédérations ont d'ores et déjà annoncé vouloir renoncer à leur part, toutes ne peuvent pas se le permettre et l'État doit prendre ses responsabilités pour accompagner et aider les acteurs. La reprise de la pratique sera difficile, nous le savons tous, mais cette crise sanitaire a également fait émerger une pratique libre ou digitale renforcée. À une époque où les individus sont demandeurs d'une pratique plus simple et sans contrainte, le développement de ce type d'activité, qui passe notamment par la digitalisation des organisations sportives, est un enjeu déterminant. Si certaines fédérations ont d'ores et déjà entamé un véritable travail sur le sujet, il est indispensable de renforcer le soutien de l'État à ces évolutions rapides. Or l'effort annoncé par le plan de relance n'est pas à la hauteur. Aussi, madame la ministre, que comptez-vous faire concrètement pour soutenir les clubs et associations lors de la reprise de la pratique ?

tandis que le sport amateur connaît une forte diminution du nombre de ses adhérents et, surtout, de ses bénévoles. Pourtant, le sport est plus que jamais indispensable pour améliorer la santé physique et mentale des Français. Nos habitudes sont bouleversées par les confinements et couvre-feux successifs. La sédentarité s'installe dans nos vies avec le télétravail. Dans un tel contexte, à trois ans des jeux Olympiques, ce débat sur l'activité et la popularité de la pratique sportive arrive à point nommé. Il s'agit d'une question essentielle, tant la pratique sportive est un facteur déterminant de santé publique, d'intégration et de cohésion sociale. Le premier objectif de la politique publique du sport, pilotée par l'État dans le cadre de la nouvelle Agence nationale du sport, devrait être l'accessibilité des lieux sportifs pour tous et la promotion du sport au quotidien.

Pour lutter contre la sédentarisation, il nous faut nécessairement renforcer la pratique sportive à l'école, d'autant plus que l'exercice physique améliore sensiblement les résultats scolaires. Or, sur les trois heures hebdomadaires de sport dispensées dans les écoles, la Cour des comptes observe que seule la moitié est effectivement consacrée à la pratique sportive. Et que dire de l'apprentissage de la natation, qui souffre d'un manque de structures ? initiatives intéressantes sont menées à l'étranger, notamment en Finlande. Favorisons les initiatives locales pour diffuser une culture du sport dès le plus jeune âge, dans le cadre scolaire ou périscolaire, et gardons à l'esprit que les temps extrascolaires sont la plupart du temps consacrés à des activités sédentaires.

Nous pourrions utilement l'intégrer dans notre politique de prévention des affections et maladies professionnelles. Il me semble que les prochains débats sur la proposition de loi pour renforcer la prévention en santé au travail seront bénéfiques à ce sujet.

Nous devons également réfléchir à l'accessibilité de ces infrastructures pour les enfants scolarisés en famille. Le sport étant parfois le meilleur des remèdes, dans le prochain projet de loi de financement de la sécurité sociale, nous ne pourrons faire l'économie d'une réflexion sur la prise en charge par la solidarité nationale de séances d'activité sportive dans le traitement des affections de longue durée. Une expérimentation pourrait être menée à ce sujet.

en lien avec les éducateurs sportifs. Nous devons encourager ces initiatives, tout en renforçant notre vigilance pour prévenir les phénomènes de radicalisation, qui s'étendent bien au-delà de l'univers carcéral et touchent le monde du sport à bien des niveaux.

démontrer. Pour reprendre les recommandations du Conseil d'État, promouvoir la pratique du sport pour tous nécessite avant tout d'instaurer un cadre sécurisé et d'étendre les contrôles réalisés par les services de l'État aux éducateurs sportifs. Pour conclure, je souligne que la politique du sport irrigue l'ensemble de l'action publique, de la santé à la cohésion nationale. Les prochaines échéances législatives seront autant d'occasions de renforcer l'accès au sport pour tous dans les meilleures conditions possible. Avant d'être la recherche de performances et de victoires, le sport est avant tout une école de la volonté, de la confiance et du vivre ensemble. Pour toutes ces raisons, nous espérons que la reprise des activités sportives en intérieur est imminente, avec des protocoles sanitaires adaptés aux différentes pratiques. Nous serons particulièrement attentifs à leur développement dans le cadre scolaire. Il faut aimer le sport et surtout le faire vivre

Dans ce monde, le sport, notamment le sport-loisir, le sport-santé, le sport populaire, doit avoir une place centrale. Dès le premier confinement, l'activité physique, même extrêmement contrainte, a souvent été le seul moment de liberté. Beaucoup ont enfilé leurs baskets pour s'évader, se libérer, y compris dans le kilomètre autorisé. Après le premier confinement, le club Vélo et Territoires a constaté une hausse de près de 28 % de la pratique du vélo par rapport à 2019. Il s'agit là d'une tendance profonde, mais fragile. Besoin de santé, besoin de vivre mieux : selon une étude de l'Université de Glasgow, réalisée en 2017 sur un échantillon de 200 000 individus, les personnes se rendant au travail à vélo voient leurs risques cardio-vasculaires ou de cancer diminuer de 40 % à 50 %. Bien entendu, cette tendance est difficilement mesurable aujourd'hui pour tous les sports. La pratique sportive en club est en chute libre, et ce pour des raisons faciles à comprendre. Dès le mois de septembre dernier, les reprises de licence étaient extrêmement variables selon les disciplines et les clubs étaient alors déjà très inquiets.

soutien aux bénévoles, le Gouvernement a déployé plusieurs mesures importantes. Ainsi, pour les clubs employeurs, aux dispositifs généraux de chômage partiel et d'allégement de cotisations viennent s'ajouter des mesures spécifiques pour l'économie sociale et solidaire en général, et pour le sport en particulier. éducation populaire, supplémentaires ou à l'aide annoncée pour la rénovation des équipements sportifs ; cela va dans le bon sens. Hélas, madame la ministre, comme dans beaucoup de domaines, dès que votre gouvernement fait un pas en avant dans la bonne direction, celui-ci est quasiment immédiatement remis en cause par un recul majeur.

ainsi que plusieurs nouvelles restrictions, notamment dans la mise à disposition des équipements. Dans un contexte de crise sanitaire où les associations sportives sont presque toutes à l'arrêt, où leurs dirigeants se démènent chaque jour pour la survie de leur structure, où les vocations des bénévoles s'amenuisent, alors que la vivacité du secteur sera la clé de la sortie de crise, le Gouvernement préfère ajouter à toutes ces difficultés des obligations aberrantes, jetant ainsi une suspicion détestable sur l'ensemble du monde sportif et associatif. En ce qui concerne l'éducation, là aussi, beaucoup reste à faire. Je le répète, l'aspiration à un mieux-être physique recouvre de nombreuses réalités, notamment dans le domaine des déplacements. La pratique du vélo nous semble ainsi particulièrement représentative de cette nouvelle réalité. Il suffit de se promener dans les artères des grandes villes ou sur les véloroutes le week-end pour le constater : jamais autant de vélos n'ont parcouru nos villes et nos campagnes. d'un moyen de transport et d'activité physique en plein boom, qui pourrait bientôt devenir le mode de transport urbain le plus utilisé, comme c'est déjà le cas dans plusieurs pays du nord de l'Europe. Pour une réelle pratique populaire du vélo, le rôle de l'éducation nationale doit être de préparer les enfants au monde de demain. Il est ainsi logique qu'elle se saisisse de ces sujets. C'est à ce titre que la loi d'orientation des mobilités de 2019 prévoit un programme d'apprentissage du vélo pour tous, afin de permettre à chaque enfant de maîtriser, à son entrée dans les établissements du second degré, la pratique autonome et sécurisée du vélo dans l'espace public. Lors de l'examen du projet de loi de finances pour 2021, nous avons été plusieurs, de tous les bords politiques, à proposer des amendements pour prolonger dans le budget de l'État cette mesure déjà votée par le Parlement. Depuis, rien n'a bougé. Madame la ministre, à ce stade, nous vous demandons plus que des promesses. Nous demandons simplement que cette mesure soit dotée du budget qu'elle mérite, dès maintenant, d'autant que votre ministère est désormais rattaché à celui de l'éducation nationale. Pour conclure, mes chers collègues, les Écologistes appellent à une politique globale en faveur du sport pour toutes et tous, une politique qui soutient ces acteurs financièrement et qui ne jette pas une suspicion permanente sur les milliers de bénévoles qui animent le sport populaire pratiqué par des milliers de Françaises et Français. Redonnons-leur des libertés, des marges de manoeuvre. Nous militons en faveur d'une politique inclusive dès le plus jeune âge et dotée d'un budget réel pour accompagner les changements profonds de notre société. La parole

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, parce qu'il recouvre une large variété de disciplines, qu'il peut être pratiqué en intérieur ou en extérieur, individuellement ou collectivement, en amateur ou en professionnel, le sport est peut-être le secteur dont on entend le moins parler depuis le 17 mars 2020. Pourtant, le sport traverse la crise la plus importante de son histoire. Depuis un peu plus d'un an, la pandémie de la covid-19 a bouleversé la vie des sportifs, en particulier celle des amateurs. Habituellement rythmée par l'organisation de plusieurs entraînements en semaine et de compétitions le week-end, la vie sportive ne peut plus se dérouler comme avant. Nous le déplorons tous. Face à l'impossibilité de se rendre dans leurs lieux de pratique habituels et face à l'arrêt des compétitions, les 18 millions de licenciés sportifs n'ont pas tous renouvelé leur licence lors du changement de saison. La perte de licenciés est estimée à 25 %, ce qui a pour conséquence la remise en cause de l'équilibre financier des associations sportives, les adhésions représentant une part importante des recettes,

Face à cette situation, ces bénévoles et ces dirigeants sportifs continuent à se mobiliser pour garder le contact avec leurs adhérents grâce aux visioconférences ou aux réseaux sociaux. Ils font aussi preuve d'innovation pour extérioriser leurs activités sportives. Les collectivités locales ne sont pas en reste pour aider leurs clubs et associations sportives. Le conseil départemental de l'Yonne, où je siège, a ainsi voté jeudi dernier un budget de plus de 2 millions d'euros en faveur du sport. Alors que notre pays continue à être dans la tempête de la covid-19, il est plus que jamais nécessaire de donner des perspectives de reprise aux sportifs amateurs et à leurs clubs, de réfléchir à la place que nous souhaitons donner au sport de demain dans notre société et à la manière dont nous souhaitons l'ouvrir au plus grand nombre. Avec la crise de la covid-19 et les confinements, l'activité sportive est apparue comme essentielle. Ce n'est pas un hasard si, parmi les mesures renforcées annoncées le 18 mars dernier par le Premier ministre pour freiner la troisième vague, figurent la possibilité de se déplacer dans un rayon de 10 kilomètres pour faire du sport, sans limitation de temps, la reprise normale de l'éducation physique et sportive sur le temps scolaire, ainsi que le maintien des activités extrascolaires en plein air pour les mineurs. Vecteur de lien social, la pratique du sport est bonne pour le physique et le moral. Avec la crise sanitaire et la progression de la sédentarité, la nécessité de rester actif est devenue une évidence pour demeurer en bonne santé. Pour bâtir le sport de demain, nous devons continuer à faire preuve d'agilité et à innover tout au long de cette crise. Pour cela, il est nécessaire que les associations sportives puissent continuer à bénéficier du soutien de l'État. Il faut le reconnaître : même si ce n'est jamais assez, le monde sportif en France est soutenu comme nulle part ailleurs dans le monde. Au-delà du plan de relance, de son volet relatif au sport, doté de 120 millions d'euros, et du déploiement du Pass'Sport en 2021, il faut continuer à lever les freins pour permettre une pratique sportive populaire et accessible à tous, mais aussi faire de la France une véritable nation sportive, comme le Président de la République s'y Cet objectif ne pourra pas être atteint sans l'aide des collectivités locales. Je le dis par expérience, en tant qu'ancienne maire adjointe de la ville de Migennes, dans l'Yonne, chargée des sports pendant treize ans. L'accueil de la Coupe du monde de rugby en 2023, puis des jeux Olympiques et Paralympiques en 2024, constitue de véritables occasions à saisir pour donner un nouveau souffle au monde sportif local. Nos territoires l'ont bien compris. Ces événements permettront de fédérer toutes les énergies locales autour d'actions variées et festives. Labélisée « Terre de Jeux 2024 » en 2019, l'Yonne a ainsi décidé récemment d'accentuer son engagement pour se positionner en tant que terre de jeux et d'accueil. Libérer les énergies sportives aura un impact positif pour nos territoires, mais aussi pour la France entière, dans le cadre de la relance. Aussi, madame la ministre, je souhaite savoir de quelle manière vous comptez encourager et amplifier la mobilisation des collectivités locales et des acteurs locaux dans le domaine du sport, dans la perspective de ces événements sportifs internationaux, et donner ainsi à nos sportifs amateurs de nouvelles perspectives positives et résolument tournées vers un avenir meilleur. La

La crise liée à la covid-19 rythme nos vies depuis plus d'un an maintenant. Pour tenter de contenir la propagation du virus, des mesures drastiques ont été mises en oeuvre. Elles ont eu des conséquences dramatiques pour nombre d'acteurs économiques, culturels ou associatifs sur l'ensemble de notre territoire. Le monde sportif a ainsi été lourdement touché. On ne compte plus le nombre d'événements annulés, reportés ou restreints au strict minimum, les championnats stoppés, qui s'ajoutent à la fermeture des lieux de rassemblement : les salles de sport, les stades, les gymnases, les piscines. Si rien n'est fait rapidement, les difficultés pourraient perdurer bien après la réouverture des infrastructures accueillant du public. Nombreuses sont les associations sportives qui font face à une évaporation du nombre de leurs licenciés et à des situations financières compliquées engendrées par le manque d'événements. Leurs adhérents, notamment les plus jeunes, les ont financées par une adhésion ou l'acquisition d'une licence, mais sans qu'aucune compétition soit organisée. Aujourd'hui, sans aucune assurance de reprise des championnats, tous ces amateurs sont dans l'expectative ; ils ne s'acquitteront pas forcément d'une nouvelle adhésion à leur club de sport. mises en difficulté par le manque de bénévoles, les associations sportives redoutent aujourd'hui des défections d'adhérents en grand nombre. Comme un problème ne vient jamais seul, l'absence de manifestations, source de recettes, et de compétitions auront aussi pour effet de faire baisser les ressources provenant des sponsors, qui peuvent représenter une part importante de la trésorerie des clubs amateurs. Les associations sportives redoutent également une chute importante du nombre de licenciés, ce qui aurait pour conséquence de mettre à mal bon nombre de championnats, notamment pour les sports d'équipe. existe aussi que les adhérents demandent un remboursement de leur cotisation. Au vu de l'ensemble de ces difficultés, le risque n'est pas nul qu'un grand nombre de ces structures ne puissent y faire face et disparaissent.

Pour qu'un retour des championnats amateurs soit possible, au-delà de l'amélioration sanitaire attendue, il faut être en mesure d'agir sur le coût de l'adhésion annuelle des licenciés. Plusieurs pistes sont à l'étude. Parmi elles, on peut citer le travail autour du dispositif Pass'Sport, qui pourrait apporter une aide à la prise en charge des licences sportives de 1,8 million de jeunes, à hauteur de 50 à 80 euros ; cela va évidemment dans le bon sens. S'assurer que la pratique du sport soit accessible à tous est d'autant plus primordial que bon nombre de jeunes basculent dans la précarité du fait de la crise. D'autres actions doivent certainement être envisagées. Dans cette perspective, et toujours afin de limiter le coût des licences et de favoriser la trésorerie des associations, pourrait-on réfléchir à un crédit d'impôt sur les frais d'adhésion ou à une déduction fiscale supplémentaire pour les dons aux associations ?

mais cela ajoute de la confusion à la confusion- c'est malheureusement une constante dans la gestion de la crise par ce gouvernement -, d'autant qu'en sens inverse, il y a quelques semaines à peine, l'interdiction de la pratique d'activités en salle avait été annoncée sans préavis, ce qui a par exemple affecté la danse. En dépit des efforts financiers des clubs pour se conformer à la réglementation sanitaire, de leur réactivité pour adapter la pratique aux nouvelles règles encadrant les lieux et les publics autorisés, et de leur capacité à démontrer leur sérieux dans la lutte contre la propagation du virus dans le milieu du sport amateur, le risque est grand de voir de plus en plus de personnes s'éloigner du sport. Déjà plus de 30 % des licenciés semblent se détourner de leurs clubs. C'est pourquoi il y a aujourd'hui unanimité pour réclamer le droit de pratiquer son sport favori. Jason Lorcher, ancien hockeyeur de haut niveau à Rouen, a ainsi lancé une pétition, voilà quelques jours. Les « sportifs en détresse » qu'il a rassemblés sont aujourd'hui plus de 30 000 à témoigner des méfaits de l'interruption de l'activité sportive amateurs, enfants, jeunes ou adultes, bénévoles ou dirigeants de clubs, tous expriment leur besoin vital de renouer avec la pratique sportive. Du point de vue de la santé, chacun sait ici combien l'activité sportive est importante pour la prévention, y compris maintenant, face au covid-19. La rupture de la pratique risque aussi de créer de nouvelles problématiques de cohésion sociale. De l'avis des professionnels de santé, les conséquences de cette interruption peuvent en effet être graves sur le bien-être, mais également sur l'équilibre psychologique ou psychique

terme, d'avoir des conséquences sur le sport de haut niveau, en asséchant le vivier dans lequel l'élite sportive puise ses ressources. Nous avons tous plaisir à regarder de grandes compétitions internationales, de beaux matchs de sport professionnel, mais ceux-ci prennent sens parce qu'ils s'appuient sur un sport amateur et populaire : ils le font rayonner, mais la réciproque est tout aussi vraie. Comment comprendre, dès lors, qu'aujourd'hui même, il y a quelques heures, les compétitions départementales et régionales de football aient été stoppées par la Fédération française de football, alors même que débutent les éliminatoires de la Coupe du monde de 2022 ?

Le Pass'Sport est un outil qui peut contribuer à lever les obstacles financiers pour tous ceux qui, dans le contexte de crise sociale actuelle, auront des difficultés à payer leur licence. Nombre de collectivités auront à coeur d'y participer. N'oublions pas cependant qu'elles aussi sont lourdement affectées, financièrement, par la crise sanitaire et toutes ses conséquences ! Il faut le prendre en compte. Il faut que les financements de l'État soient au rendez-vous si nous voulons que le Pass'Sport suscite véritablement la reprise de licences par le plus grand nombre. connaissons doit être l'occasion de revoir en profondeur le financement de notre modèle sportif et de porter un plan ambitieux en matière de sport. Je salue à mon tour l'ensemble des propositions qui ont été émises sur toutes les travées de notre assemblée à l'occasion de ce débat. Vous avez là, madame la ministre, des propositions à la fois

Le sport est encore un enjeu populaire : on compte 10 millions de licenciés dans les différentes fédérations sportives ; deux Français sur trois pratiquent toutes les semaines une activité sportive régulière.

Aucun autre événement ou mouvement social populaire ne peut rassembler autant de personnes aussi régulièrement

des protocoles spécifiques puissent être expérimentés dans nos collectivités, nos départements et nos territoires. C'est un enjeu majeur. Je terminerai mon propos par une citation de Jean Giraudoux : « Il y a des épidémies de tout ordre ; ; le goût du sport est une épidémie de santé. » Puisse cette épidémie de santé durer le plus longtemps possible !

le monde sportif souffre depuis près d'un an. À ce jour, il n'a aucune perspective de reprise ; seuls les clubs professionnels sont pleinement autorisés à pratiquer avec contact et à prendre part à des compétitions à huis clos. Ce n'est pas idéal, mais c'est adapté et proportionné à la situation sanitaire. En revanche, le sport amateur, la grande majorité des clubs semi-professionnels et les salles de sport restent sur la touche. Les clubs semi-professionnels et amateurs sont tous soumis au même régime, qu'ils prennent ou non part à des compétitions nationales ou continentales. D'après les consignes qu'ils ont reçues de la part de la direction des sports, seuls les clubs comptant plus de 70 % de sportifs professionnels peuvent s'entraîner sans distanciation et prendre part à des compétitions. Ce critère n'est absolument pas adapté à la réalité du monde sportif et met de côté un grand nombre de clubs qui évoluent dans des compétitions de haut niveau. Madame la ministre, je vous ai envoyé un courrier pour vous alerter de la situation dans laquelle se trouvent ces clubs qui rassemblent à la fois des sportifs de haut niveau, qui sont autorisés à s'entraîner avec contact, des sportifs amateurs, qui ne peuvent s'entraîner que sans contact et en dehors du couvre-feu. En raison de ce critère de 70 %, la plupart de ces clubs ne peuvent pas prendre part à des compétitions ni s'entraîner de façon adaptée pour celles-ci. Je vous ai alors proposé de fixer différemment les critères, en autorisant les compétitions et les entraînements sans distanciation uniquement pour les clubs évoluant à l'échelle nationale ou européenne. Ceux qui ne prennent part qu'à des compétitions départementales ou régionales n'y seraient pas autorisés. Dans votre courrier de réponse, vous m'avez indiqué que permettre la reprise des entraînements avec contact pour l'ensemble du sport amateur n'était pas adapté à la situation sanitaire. Il ne s'agit absolument pas de permettre une reprise pour tous, cette demande concerne les seuls clubs prenant part à des compétitions de haut niveau et ayant de ce fait des budgets importants que les aides actuelles ne peuvent compenser. Cette règle des 70 % a des conséquences désastreuses pour les clubs. La majorité des fédérations ont dû annuler les championnats de France et plusieurs devront rompre les engagements qu'ils avaient pris dans le cadre des championnats européens. Plusieurs clubs voient leurs membres les quitter pour d'autres, situés dans des pays étrangers où les compétitions amateurs ou semi-professionnelles sont autorisées, tels que la Suisse, l'Italie, la Finlande, l'Espagne ou encore l'Allemagne. Malheureusement, il est déjà trop tard pour rattraper cette situation. Il faut donc maintenant tout miser sur la saison prochaine. Les clubs sont conscients de la situation sanitaire et leurs revendications sont proportionnées à celle-ci. D'une part, ils souhaitent une reprise des sports collectifs avec contact avant l'été, en priorité pour les jeunes. Cela leur permettra de sécuriser leurs inscriptions pour la rentrée de septembre si d'ici à l'été la situation sanitaire n'est pas suffisamment stabilisée pour permettre une reprise du sport pour tous, les clubs souhaitent que le sport sans distanciation et les compétitions soient possibles uniquement pour ceux d'entre eux qui évoluent dans des compétitions nationales et européennes, pour les jeunes comme pour les adultes.

Vous engagez-vous de ce fait à ne pas laisser le sport collectif à l'abandon et à étudier leurs propositions raisonnables et sensées ? Enfin, j'en viens à la situation des salles de sport. Déjà fermées durant le premier confinement, elles le sont de nouveau depuis le mois d'octobre dernier. Elles sont aidées au titre du fonds de solidarité, mais celles qui enregistrent moins d'un million d'euros de chiffres d'affaires par mois ne sont pas éligibles à l'indemnisation de leurs charges fixes. Cela changera au début du mois d'avril prochain, mais seuls les mois de janvier, février et mars seront indemnisés de façon rétroactive, alors que les charges sont supportées depuis de nombreux mois. Plus de 300 salles ont déjà déposé le bilan et il a fallu plus d'un an pour que leurs alertes soient entendues. Quel gâchis ! Le sport participe pourtant à la lutte contre la pandémie, puisque les personnes en bonne santé et pratiquant une activité physique régulière ont moins de chances de souffrir d'une forme grave de la covid-19. La plupart des études prouvent en outre que, si le sport sans masque en milieu fermé favorise la propagation du virus, une pratique sportive en intérieur avec masque, distanciation et aération présente très peu de risques. Si l'interdiction d'ouverture peut se comprendre dans les départements confinés ou en surveillance, elle est loin d'être proportionnée dans ceux où les taux d'incidence sont bas. Le Gouvernement a commencé à territorialiser les mesures de lutte contre l'épidémie, mais il faut aller plus loin et faire de même pour l'ouverture des salles de sport. Des critères supplémentaires peuvent être fixés, tels qu'une surface suffisante pour pratiquer la distanciation et des moyens d'aérer la salle. Interdire à toutes les salles d'ouvrir sur tout le territoire n'est pas proportionné.

Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, mes chers collègues, qui font écho aux témoignages des licenciés que j'ai rencontrés, évoquant les risques qui pèsent sur leurs fédérations et leurs clubs, une évidence apparaît : le rôle du sport dans nos sociétés.

Plutôt que l'interdiction brutale, l'État aurait dû et pu instaurer avec eux un protocole adapté à la crise. En effet, non seulement aucun cluster n'est apparu dans ces établissements, mais des mécanismes d'identification à l'entrée permettent de tracer l'heure d'arrivée des adhérents et d'identifier les personnes croisées. Plus généralement, les gérants et les responsables associatifs qui assurent le fonctionnement des équipements sportifs connaissent mieux que quiconque les gestes et les déplacements qui y sont pratiqués. ils n'ont pas été consultés, alors qu'ils auraient pu être des auxiliaires précieux pour éliminer le virus sans détruire le sport. Il faudra s'en souvenir demain. Il faudra aller chercher des solutions innovantes.

Devons-nous pour autant continuer à renoncer totalement à nos activités sportives, avec les conséquences que chacun a déplorées ici ? Non ! Concentrons plutôt nos efforts sur la diffusion de masques adaptés à un large éventail de disciplines, notamment les sports collectifs. Une entreprise ardéchoise, Chamatex, développe justement de tels masques, qui n'entravent pas la respiration et permettent une mobilité impensable avec les modèles basiques. Soutenons-la ! ! Encourageons ainsi partout le génie du pragmatisme, ce qui sifflera la fin de cet interminable arrêt de jeu. Au-delà de cette épidémie dont nous finirons par venir à bout, le temps est déjà venu de réfléchir aux crises de demain. Je pense à notre future capacité à passer, en cas de nouvelle alerte épidémique et dans un délai minimal, à une organisation adaptée à nos pratiques sportives, individuelles ou collectives. Les orateurs précédents l'ont souligné : faute d'anticipation, nous découvrons brutalement les conséquences de la privation de sport sur la population. Il faut donc, madame la ministre, que vos services travaillent dès à présent sur un qui serait directement efficient en cas de nouvelle crise. Il permettrait aux associatifs, aux professionnels, aux élus et aux sportifs de basculer immédiatement dans un fonctionnement de crise, avec des règles du jeu connues, puisque déjà définies en amont. Les acteurs du secteur, comme le collectif événementiel sportif Outdoor, très actif dans mon département, proposent des expérimentations encadrées pour sauver des événements sportifs grand public en plein air. Accompagnons-les ! En 2020, nous avons été surpris et désemparés. Aujourd'hui, nous devons prévenir un futur épisode pandémique avec l'état d'esprit des athlètes de haut niveau, c'est-à-dire en nous jurant d'être prêts le jour de l'épreuve. Pour paraphraser une devise célèbre, je dirais que nous devons passer à ce format adapté plus vite, avec des niveaux de maintien de la pratique plus hauts, et que nous en sortirons plus forts. Madame la ministre, à vous qui avez en votre temps prononcé le serment olympique, il appartient de prendre ce soir devant nous ce nouvel engagement ! Mes chers

je suis arrivée à la tête de ce ministère, une réforme était déjà en cours, engagée par Laura Flessel, dont l'ambition était de nouer une relation différente avec le mouvement sportif.

également question d'un lien plus fort entre l'instance fédérale, les clubs et les adhérents au travers des modalités de vote au sein des instances dirigeantes des fédérations.

Enfin, le titre III traite du modèle économique que vous avez évoqué à plusieurs reprises ce soir. Comment protéger le modèle économique du sport en France ?

je suis très attachée à la régulation du modèle économique du sport. Je suis également très attachée à la solidarité entre le sport amateur et le sport professionnel. Ayant été moi-même sportive de haut niveau, je connais le parcours et le circuit que suit tout

en collaboration, encore une fois, avec les territoires, les mouvements sportifs et toutes les entreprises, qui sont aussi convaincues que le sport est essentiel au bien-être physique et psychologique des Français.